La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local

vous évoquez l’idée que puissent être créées trois enveloppes – une pour les maires, une pour les adjoints, une pour les conseillers délégués et conseillers municipaux – et vous sollicitez mon avis

Nous proposons donc que l’indemnité du maire soit sacralisée, c’est à dire qu’elle ne soit pas discutable. C’est clair ! Deuxièmement, nous proposons qu’il en soit de même pour les adjoints. Troisièmement, mes chers collègues, nous sommes tous ici des élus locaux et nous n’arrêtons pas de dire qu’il faut permettre aux élus locaux de s’administrer et de s’adapter à des différenciations.

rapporteur. Je rappelle que cette proposition de loi a été construite collectivement, que nous avons essayé, pour chacune des mesures, de trouver celle qui nous semblait la plus opérationnelle, la plus concrète, pour traiter

à l’article 2. Le présent amendement vise tout simplement à rendre opérationnel le principe selon lequel les indemnités de fonction des exécutifs locaux sont fixées, par défaut, à leur maximum légal. Bien entendu,

du débat politique des élections municipales l’enveloppe globale des indemnités et des frais de fonction.

M. Laurent Somon. Cet amendement tend à supprimer l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, afin de garantir l’indemnisation des conseillers simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires. Dans le contexte actuel, l’enveloppe indemnitaire globale, calculée en fonction du nombre maximum théorique d’adjoints, ne laisserait aucune marge de manœuvre pour indemniser les conseillers municipaux simples ou délégués lorsque le nombre maximum d’adjoints a été élu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Vous proposez de supprimer le seuil qui réserve la faculté de moduler les indemnités de fonctions des élus selon leur assiduité dans les communes de plus de 50 000 habitants.

ouvrant droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de sorte que tout élu local, même non membre d’un exécutif, puisse bénéficier d’une indemnité de chômage lorsqu’il quitte son mandat pour cause de non réélection.

Or des élus se sont vu répondre par leur administration que, si le crédit d’heures n’est pas rémunéré par l’employeur, la période concernée ne donnera pas lieu à cotisations et ne sera pas prise en compte, faute de texte législatif ou réglementaire le prévoyant explicitement au titre des droits à pension de l’État.

sur un point important. La plupart des élus locaux investissent leur temps et leur énergie sans compter les heures, parfois au détriment de leur vie professionnelle et familiale. Conjointement, on observe un véritable risque de désengagement des citoyens, notamment des plus jeunes, dans la prise de responsabilités politiques, ce qui, par voie de conséquence, fait pâtir notre système démocratique et sa représentativité. La possibilité de bonifier la retraite des élus locaux sous la forme de l’attribution de trimestres supplémentaires, telle qu’elle est proposée par la commission, est une excellente idée.

que la ruralité connaît ces dernières années et dont la crise agricole est le symptôme. En 2020, nous avions voté la revalorisation des retraites agricoles de manière unanime sur ces travées. Or, près de quatre ans plus tard, la situation est loin de

Quel est l’avis de la commission ?

pour les raisons qui ont déjà été avancées. Il nous semble absolument fondamental que l’engagement des élus soit reconnu au moment de leur retraite.

est à Mme le rapporteur. Cet amendement vise à élargir la bonification de trimestres de retraite à tous les élus municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions.

qui ne disposent de presque aucun mécanisme efficace et lisible. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport de clarification, d’évaluation et de proposition relatif au dispositif

de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés en raison de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime au titre de mandats locaux en cours ou échus.

par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à des difficultés qui n’ont pour effet que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à la pension professionnelle à laquelle ils ont normalement droit. À titre d’exemple, à ce jour, cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus qui sont par ailleurs avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leur indemnité ou à démissionner, et cela malgré les évolutions issues de la dernière réforme des retraites.

En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal en raison de la prise en compte de la pension Ircantec. Il apparaît donc aujourd’hui plus que nécessaire de sanctuariser dans la loi la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension par d’autres régimes de retraite. Tel est l’objet de cet amendement.

n° 44 rectifié. Monsieur le sénateur Roiron, vous souhaitez limiter les interférences entre l’Ircantec, auquel sont affiliés les élus locaux, et leurs régimes professionnels. Cet objectif est partagé par le Gouvernement, qui a déjà pris différentes mesures, afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local. En ce qui concerne les minima de pension, la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l’Ircantec, afin de permettre aux élus concernés de bénéficier des minima de pension et des majorations de pension de réversion. Néanmoins, le calcul de ces minima peut faire l’objet d’un écrêtement dont le plafond s’apprécie en prenant en compte l’ensemble des pensions de l’assuré, de base et complémentaires, françaises

a sanctuarisé la possibilité pour les élus d’ouvrir des droits à l’Ircantec après la liquidation de leur pension. Néanmoins, des difficultés persistent, notamment au regard de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l’ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi retraite libéralisé. Cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours, du fait de droits demeurant ouverts à l’Ircantec. En effet, une lettre ministérielle de 1996 prévoit que les élus locaux ne peuvent pas liquider leurs droits à l’Ircantec avant la fin de leur mandat, alors qu’une telle liquidation permettrait à un élu de satisfaire à la condition de subsidiarité. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à supprimer cette lettre ministérielle de 1996, afin qu’un élu local puisse justifier de la condition de subsidiarité exigée en liquidant ses droits à l’Ircantec sans avoir à interrompre son mandat ou à en attendre la fin. Par ailleurs, le Gouvernement prévoit de déposer un amendement permettant de préciser les règles d’ouverture, de constitution et de liquidation des droits à l’Ircantec pour les élus locaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’avez compris, nous sommes défavorables à cet amendement ;

Ils ont ainsi constitué des droits auprès de ces régimes extra légaux de retraite par répartition, portés juridiquement par de simples associations de loi 1901. Le législateur a entendu mieux encadrer ces pratiques, en définissant un régime unifié de retraite pour les élus, l’Ircantec, tout en mettant en extinction les régimes existants, dans l’article 32 de la loi du 3 février 1992 Les droits acquis au sein de ces régimes ont en outre été préservés : les pensions liquidées tout comme les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés. De plus, les élus en fonction, ou ayant déjà acquis des droits dans ces régimes avant le 30 mars 1992, ont été autorisés à continuer à cotiser, la collectivité devant alors apporter une contribution égale à celle de l’élu. L’extinction progressive de ces régimes entraîne néanmoins, pour les associations concernées, des difficultés croissantes pour assurer leur gouvernance, leur fonctionnement et leur financement. C’est pourquoi plusieurs départements ont transféré la gestion de ces régimes historiques à un acteur tiers, la Caisse des dépôts et consignations.

Il convient donc d’en clarifier la possibilité dans la loi. Tel est l’objet de cet amendement, au bénéfice des élus concernés.

la pension d’invalidité, ou de bourses étudiantes sur critères sociaux, les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte, au moins en partie, dans le montant des ressources qui sert de base au calcul. Ainsi,

en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général. La

par le Gouvernement au Parlement d’un rapport relatif aux coûts qui pèsent sur les communes, liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État, dans de nombreux domaines : publication et exécution des lois, règlements, charges d’officier de police judiciaire ou d’état civil,

prévoir un rapport relatif au coût des compétences exercées au nom de l’État avant le 30 juin 2025. Je rappelle tout d’abord que la loi de finances pour 2024 vient de procéder à une revalorisation de la DPEL de 15 millions d’euros. de 15 millions d’euros. En 2019, la DPEL était à 65 millions d’euros ; dans le PLF pour 2024, elle est à 130 millions d’euros. Cette revalorisation vise à couvrir, tout d’abord, une meilleure prise en compte du coût de la protection fonctionnelle des élus pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants, qui deviennent éligibles à la majoration dédiée de la DPEL, jusqu’alors réservée aux seules communes de moins de 3 500 habitants

mais j’ai plaisir à vous le rappeler. Les communes de moins de 3 500 habitants perçoivent en outre d’ores et déjà une fraction de DPEL pour le financement de la garde d’enfants et de la protection fonctionnelle. Au demeurant, le relèvement du seuil d’éligibilité de la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants aurait pour conséquence d’y rendre éligibles près de 32 000 communes,

par les maires de missions de l’État, il convient de rappeler qu’il s’agit de missions historiques, pour la plupart d’entre elles, assurées depuis la création de la commune, avant même la décentralisation, et qui ne sauraient donc bénéficier du régime juridique des compensations liées au transfert de compétences. Compte tenu de ces éléments, je propose la suppression de l’article 4. Quel

Cette dotation vise principalement à compenser les dépenses obligatoires résultant des dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Elle est prélevée sur les recettes de l’État pour assurer le bon fonctionnement de la démocratie locale. Ces difficultés que connaissent de plus en plus de petites communes sont de votre responsabilité, madame la ministre, car elles résultent

Permettez moi toutefois, madame la ministre, d’attirer votre attention sur la nécessité d’augmenter significativement ces dotations et d’en simplifier l’accès, pour qu’elles puissent bénéficier au plus grand nombre de nos communes, en particulier aux plus petites d’entre elles, et cela dès la prochaine loi de finances. Quel

les démissions de maires – 1 078 – et de conseillers municipaux – 29 214 –, s’accélèrent par rapport au mandat 2014 2020. seraient en augmentation de près de 30 %. Risques d’incivilités ou d’agressions, sentiment que la charge est trop lourde, difficultés à concilier leur mandat avec leur vie professionnelle et personnelle : le mal être des élus locaux est bien identifié aujourd’hui. Pour faire face aux violences psychologiques que subissent les élus, le Gouvernement a certes mis en place un numéro vert au mois de novembre dernier, mais il n’existe à ce jour aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus.

déléguée. Cet amendement vise à compléter les dispositifs de remboursement de frais de transport prévus pour les communes et pour les EPCI. L’article 5 tend notamment à rendre obligatoire le remboursement des frais de transport et de séjour engagés par les élus locaux lorsqu’ils représentent leurs collectivités. Il prévoit en outre, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une compensation par l’État des remboursements des frais de déplacement. déplacement. Les élus ont déjà droit au remboursement de frais de transport, sous réserve des conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, à savoir un critère matériel lié à la nature de la réunion et un critère géographique pour les élus municipaux et d’établissements publics de coopération intercommunale.

prévoir le remboursement des frais de transport engagés par les élus municipaux pour se rendre aux réunions et séances qui ont lieu sur le territoire de la commune, ce qui couvrira certaines difficultés de remboursement rencontrées par les élus, par exemple pour leurs déplacements

en prévoyant, d’une part, que les modalités de remboursement soient fixées par délibération des assemblées et, d’autre part, que les notes et les justificatifs de frais puissent être communiqués Le Conseil d’État, dans une décision du 8 février 2023, a jugé qu’un maire ne pouvait pas refuser de transmettre ses notes de frais de restauration et de représentation à tout citoyen qui en ferait la demande, puisqu’il s’agissait de documents administratifs. Il est donc important, pour

en encadrant le montant des remboursements fixés par délibération en conseil départemental ou régional et en prévoyant une communication de ces documents.

aux membres du conseil territorial de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon est l’article L. 6434 5 du CGCT. Par conséquent, l’application du dispositif à Saint Pierre et Miquelon devrait être prévue à cet article. En outre, la mesure que vous proposez concerne l’extension à Saint Pierre et Miquelon de la possibilité pour le conseil territorial de voter des frais de représentation pour son président. Cette disposition portant sur les relations entre deux institutions de la collectivité, et non sur le régime indemnitaire d’un élu du conseil, elle devrait être inscrite dans une loi

en permettant aux présidents de département et de région de bénéficier du remboursement des frais de représentation. Toutefois, il ne prévoit pas expressément le bénéfice de cette faculté pour le président de l’assemblée de Guyane, le président de l’assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Le présent amendement vise donc à corriger cette

aux conseillers municipaux en déplacement professionnel loin de leur commune de continuer de participer aux réunions du conseil et donc de prendre part aux délibérations.

! Ce n’est pas une première. Je me souviens que, lorsque nous avions examiné la loi 3DS, il y avait également eu un oubli,

de l’action publique locale) qui prévoit la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux. Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, cet amendement vise à ouvrir aux bureaux des communautés de communes et des métropoles la possibilité de se réunir en visioconférence.

auprès des citoyens en les autorisant à faire figurer une cocarde tricolore sur leur véhicule.

l’utilisation de la cocarde est encadrée par l’article 50 du décret n° 89 655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Cet article dresse une liste limitative des autorités autorisées à utiliser la cocarde aux couleurs nationales sur les voitures officielles. Les élus locaux, dont les maires, ne font pas partie de cette liste et ne sont par conséquent pas autorisés à faire figurer la cocarde sur leur véhicule. L’amendement est donc irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution, son objet relevant non pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire. Sur le fond,

Toute restriction apportée à l’exercice des fonctions publiques par la définition de l’incompatibilité visée par cet amendement doit être justifiée, conformément aux exigences de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la nécessité de protéger le libre choix de l’électeur et l’indépendance de l’élu. À ce titre, le Conseil d’État a estimé, dans une décision du 17 décembre 2014, qu’en instaurant cette interdiction prévue à l’article L. 237 1 du code électoral le législateur n’a pas excédé le strict nécessaire pour protéger la liberté de choix

article prévoit de porter à vingt, contre dix actuellement, le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence dont peut bénéficier un candidat à une élection locale au titre du congé électif, dispositif qui a été étendu aux candidats aux élections territoriales et provinciales en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie. Le recours à un congé électif prolongé par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques

705 316 candidats aux élections municipales qui seraient susceptibles d’accéder à vingt jours de congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période du scrutin.

Enfin, il convient de noter que la proposition de loi exclut les élections européennes en maintenant la durée du congé électif à dix jours pour ceux qui y sont candidats, alors même que la durée de la campagne électorale régie par l’article 15 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est similaire à celle prévue par l’article L. 47 A du code électoral. Cette absence d’harmonisation n’est, elle non plus, pas justifiée. Elle est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats au scrutin européen et les autres candidats, et complexifierait le droit existant. Pour ces raisons, le Gouvernement vous propose la suppression de l’article 8 de la proposition de loi. Quel

aux temps d’absence que l’employeur est tenu d’accorder à son salarié pour les cérémonies publiques, comme le prévoit l’article 9, les missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. La mention de ce mandat spécial exclut les activités courantes de l’élu. Elle permet de couvrir des opérations déterminées de façon précise et accomplies dans l’intérêt de la collectivité, par exemple une manifestation de grande ampleur ou un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité. Cette hypothèse comprend, par exemple, le cas de catastrophe naturelle. Cette notion est à la fois souple, puisqu’aucune liste n’est définie, tout en visant des opérations indispensables et inhabituelles dans l’exercice d’un mandat, ce qui permet de limiter les contraintes induites pour l’employeur. L’attribution d’un mandat spécial exige par ailleurs nécessairement une délibération, ce qui permet de justifier la nécessité de l’absence de l’élu. Un mandat spécial peut également être attribué dans des conditions d’urgence, la délibération prise à cet effet pouvant alors être postérieure à l’exécution de la mission. Cela permet à l’élu de s’absenter en cas de circonstances exceptionnelles. Ce dispositif rejoint ainsi l’objectif de l’article 9 dans sa rédaction initiale, à savoir mettre en place une procédure dérogatoire d’absence en cas de crise ou d’urgence. Le présent amendement étend ces nouvelles autorisations d’absence aux élus municipaux, départementaux et régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane et aux membres de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Il modifie en conséquence la rédaction des articles concernés et les harmonise, en complétant notamment l’article relatif aux conseillers régionaux. Le 2° reprend l’apport de la commission qui prévoit la faculté pour l’employeur de rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits et l’étend à tous les élus bénéficiant de ce dispositif. Le 3° augmente le nombre d’heures susceptibles d’être compensées par la commune pour les élus municipaux qui exercent une activité professionnelle, salariée ou non, qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction. En effet, les périodes de temps garanties aux élus locaux par le mécanisme des autorisations d’absence et du crédit d’heures ne sont pas nécessairement rémunérées par les employeurs. Elles occasionnent ainsi une perte de revenus

Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du Smic, soit 17,47 euros, ce qui fait un montant maximal brut par an de 1 257,84 euros par élu. Ce dispositif n’a pas fait l’objet de revalorisation depuis 2002, la loi du 27 février

le montant maximal brut de la compensation à 1 747 euros par élu, soit une augmentation de 39 %. Quel est l’avis de la commission ?

alerte rouge est déclenchée par le préfet, la sécurité de nos concitoyens devient une priorité. Certains membres du conseil municipal cumulent cependant leurs responsabilités avec une activité professionnelle dans le secteur privé.

Cette mesure simple tend à garantir une participation effective des membres du conseil municipal à la situation d’urgence. En leur offrant ce temps de repos, nous nous assurons que ces derniers puissent répondre de manière optimale aux enjeux de sécurité et aux mesures d’urgence, en contribuant à une gestion efficiente des crises et en démontrant leur engagement en faveur de la sécurité de la population.

Les rapporteurs, lors de l’examen du texte en commission, ont restreint cette procédure aux seuls maires et adjoints. Mais les petites communes ont besoin de l’ensemble de leurs équipes lorsqu’un événement climatique a lieu,

donner instruction aux différents développeurs de logiciel de paie de créer une nouvelle dénomination dans la catégorie des absences, permettant de renommer une absence non rémunérée en en « absence d’élu de la République » afin de matérialiser et valoriser l’engagement des salariés élus. Quel est l’avis de la commission

régional ou départemental, de suspendre son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat. Mais cette possibilité est limitée aux salariés justifiant une ancienneté minimale d’un an.